L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020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

Elle permet de soulager la trésorerie des TPE et PME des secteurs les plus touchés par la crise. Bien sûr, une telle mesure n'est pas suffisante en soi. C'est pourquoi elle doit trouver à s'intégrer dans une politique économique globale de soutien aux entreprises. L'amendement que je vous propose de voter vise à élargir ce dispositif aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui jouent un rôle essentiel dans l'économie des territoires. L'élargissement du champ d'application de cette mesure présente un double avantage d'une part, il envoie un signal positif aux dirigeants des ETI en les intégrant pleinement dans la stratégie de soutien aux entreprises ; d'autre part, il représente un coût relativement faible pour les finances publiques, compte tenu de la composition du tissu des entreprises concernées par la mesure.

compte tenu de l'obligation de fermeture administrative et de l'interruption brutale des flux touristiques. Les outre-mer ont ainsi été très fortement touchés par la crise. des initiatives ont été prises pour soutenir le secteur, mais la crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et durable. Nombreuses sont celles qui risquent de ne pas échapper au dépôt de bilan. Aussi, les dispositifs d'aide mis en place doivent perdurer encore un certain temps, afin de permettre à ces entreprises de se relever. Cet amendement, très important pour la profession, vise donc à prolonger la période d'annulation des redevances et produits de location dus au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'État et de ses établissements publics pour les CHR,

J'ajoute que l'amendement n° 35 a pour objet d'étendre la période d'exonération jusqu'à la fin de l'année 2020, ce qui nous paraît, excusez le terme, un peu exubérant, dans la mesure où nous avons calé les dispositifs d'exonération sur la période pendant laquelle l'occupation était interdite ou empêchée pour les bénéficiaires de la concession.

sur tout le territoire. Dans l'alimentaire, il accuse en moyenne des baisses de chiffre d'affaires entre 30 % et 50 %, et jusqu'à 70 % à 100 % pour les commerces et artisans non sédentaires vendant des produits manufacturés. Après l'arrêt brutal des activités des commerces ne vendant pas des produits de première nécessité, les commerces de bouche non sédentaires se sont retrouvés dans une situation instable et précaire, dans la mesure où les textes réglementaires les ont d'abord autorisés à poursuivre leur activité, avant de prévoir une nécessaire autorisation du préfet, ainsi que des mesures organisationnelles et de contrôle pour qu'ils puissent fonctionner, et ce pendant près de deux mois. Le commerce de bouche non sédentaire, composé de très petites entreprises de proximité, s'est retrouvé concurrencé par la grande distribution, laquelle a été autorisée à ouvrir par défaut et sans autorisation, contrairement aux marchés. Afin de soutenir des secteurs largement fragilisés, il convient d'aller au-delà des suspensions de la redevance au titre de l'occupation du domaine

cet amendement a pour objet de créer une dérogation afin que les activités d'avitaillement d'aéronefs et de trains exerçant sur les plateformes aéroportuaires et ferroviaires ne soient pas soumises à la définition européenne de la PME pour bénéficier de l'exonération des redevances domaniales et commerciales. De fait, la limitation des exonérations aux entreprises de moins de 250 salariés dans ce secteur n'a pas de sens, car les trois opérateurs existants sont des ETI. Par conséquent, le dispositif conservé en l'état exclurait des exonérations de redevance l'ensemble du secteur pourtant éligible au plan d'aide à la filière tourisme, et qui représente à lui seul 12 500 salariés sur le territoire français. Quel est l'avis de la commission ?

et de l'interruption brutale et totale des flux touristiques en mars. Malgré les initiatives prises par le Gouvernement pour soutenir le secteur, la crise à laquelle font face ces entreprises est profonde et vraisemblablement durable. d'une reprise d'activité lors du déconfinement, nombreuses sont celles qui risquent purement et simplement de ne pas échapper au dépôt de bilan. Les dispositifs d'aide qui ont été mis en place doivent durer dans le temps pour permettre à ces entreprises de se relever. Cet amendement, très important pour la profession, vise donc à à faire passer de trois mois à neuf mois, dans les mêmes conditions, la période d'annulation des redevances et produits de location dus au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'État et de ses établissements publics pour les entreprises du tourisme.

l'avis du Gouvernement ? D'abord, je veux rappeler la logique du Gouvernement, qui n'est pas tout à fait la même que celle de la commission. Nous avons pensé le dispositif d'exonération non pas sur la période de l'état d'urgence, mais sur la période pendant laquelle l'accès aux établissements concernés était empêché

physique d'accéder aux lieux et aux concessions, l'emporte sur la durée de l'état d'urgence sanitaire, lequel ne s'accompagne pas systématiquement d'une interdiction d'accès aux établissements concernés.

Cet amendement, déposé par mon collègue Vincent Delahaye, tend à revenir sur la création d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique, ou à un service de presse en ligne. le but de l'impôt doit rester le financement d'une action publique et non devenir le déterminant des comportements individuels. Par ailleurs, face aux conséquences économiques terribles de la pandémie de covid-19, la responsabilité impose d'établir des priorités en matière de dépenses publiques. Aussi louable

je ne suis pas certain qu'un crédit d'impôt de 50 euros pour un premier abonnement suffise à sauver la presse. C'est de la com' ! Je suis conscient du caractère quelque peu symbolique de cette mesure de saupoudrage,

la presse en ce moment, tout ce qui peut donner le sentiment d'être un début de commencement d'aide n'est pas malvenu. Autant, comme je l'ai déjà dit au précédent ministre

Mme Céline Brulin, pour explication de vote.

l'attribution de la prime covid aux structures de la petite enfance. Pendant la crise sanitaire, de nombreuses crèches ont continué d'exercer leurs missions, non sans difficultés et avec un grand mérite, notamment pour permettre aux parents soignants ou socio-éducatifs auprès des patients, personnes handicapées et âgées de poursuivre leurs activités d'aide et de soins, ainsi qu'aux parents salariés travaillant dans des secteurs essentiels, tels que la grande distribution. Il serait juste que les personnes travaillant dans les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans restés ouverts pendant la crise sanitaire bénéficient de cette prime exceptionnelle. Quel est l'avis de la commission

les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et autres établissements sociaux et médico-sociaux, pour faire face à l'épidémie de covid-19 et continuer d'apporter des services essentiels au bien-être des patients et résidents, du soin à la fourniture de repas, sans oublier le nettoyage des locaux et des chambres.

et remplissant les conditions d'une présence effective et continue dans les établissements pendant la crise sanitaire. C'est une question d'égalité pour ces personnels qui ont beaucoup oeuvré.

défavorable. Les prestataires privés qui interviennent dans le champ médico-social ne sont pas des salariés d'un établissement médico-social et, en cela, n'entrent pas dans le champ de la prime covid.

et qui est ouverte aux entreprises du secteur privé, dépend- vous ne l'avez pas dit, mais je le précise -de la volonté et de la décision du chef d'entreprise, de la même manière d'ailleurs que la prime qui est ouverte aux agents de la fonction publique territoriale dépend,

fait le choix d'une augmentation de salaire pour l'ensemble des soignants et des personnels médico-sociaux. Très bien

en tête. Dans la mesure où l'État verse une prime pour reconnaître l'engagement des salariés des groupes privés gestionnaires, pourquoi traiterait-il différemment les salariés des sous-traitants ?

de la prime au profit des employeurs médico-sociaux a été arrêté par un arrêté du ministre de la santé et des solidarités, pour que les employeurs puissent être accompagnés dans le financement de la prime. Nous avons besoin de la loi pour les exonérations de cotisations et les exonérations de fiscalité. Lorsque la prime est automatique parce qu'elle est financée sous Ondam, l'exonération est prévue. Lorsque les salariés relèvent du secteur privé ou de la fonction publique territoriale, où, je le répète, la prime est facultative et à la main des employeurs,

selon la date à laquelle ont été acquis les titres. [ ...] En effet, un contribuable qui détient des titres depuis plus de deux ans et moins de huit ans a intérêt à choisir le barème progressif et ainsi profiter des abattements.

! Nous proposons que l'abattement de 40 %, applicable aux revenus distribués par les sociétés françaises ou étrangères ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales- fiscalité

est relativement attractif et compétitif par principe, cette imposition forfaitaire est assise sur le montant brut des revenus concernés. En second lieu, je précise que l'abattement de 40 % est, lui, maintenu en cas d'option du contribuable pour l'imposition de ses revenus mobiliers suivant le barème progressif.

en cette période de crise sanitaire. Par ailleurs, cet abattement répond à une logique : il s'agit de prendre en compte le fait que les revenus distribués ont déjà été imposés à l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas la première imposition à laquelle ils sont soumis. J'ajouterai deux choses. La première, c'est que,

pas devenus fous, ne souffrent pas d'un effet collatéral de la pandémie. Ils expliquent dans leur appel : « Nous avons une dette énorme envers les gens qui travaillent en première ligne dans cette bataille globale. Des salariés essentiels sont largement sous-payés pour la charge qu'ils portent. À l'avant-garde de ce combat se trouvent nos personnels soignants, dont 70 % sont des femmes. Ils affrontent le virus mortel chaque jour, tout en assumant la plus grande responsabilité pour le travail à la maison non rémunéré. Le risque que ces personnes courageuses prennent pour prendre soin de nous nous impose d'établir un véritable nouvel engagement de solidarité avec ce qui compte vraiment. Taxez-nous

pour réduire la charge pesant sur les Français les moins riches et pour augmenter la contribution des Français les plus fortunés, pour des raisons d'équité, mais également d'équilibre financier.

ainsi que les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sur les revenus du patrimoine et la tranche marginale à 60 % que vous proposez de créer, nous aboutirions à un niveau de taxation global qui pourrait être considéré comme confiscatoire par le Conseil constitutionnel. À cet égard, M. le rapporteur général a rappelé les décisions

En France, les milliardaires ne donnent pas assez. Cette crise va propager la misère et creuser les inégalités. Je souhaiterais de leur part des paroles et des actes forts afin d'afficher leur solidarité.

% des Français sont favorables à une taxation accrue des millionnaires. Seuls 20 % la désapprouvent. En Allemagne, c'est très exactement

Cette prime reposant entièrement sur les finances des départements, son coût peut potentiellement décourager ces collectivités, et ce plus particulièrement lorsqu'elles ont été très touchées par l'épidémie.

nous sommes fidèles aussi à la doctrine de non-compensation lorsqu'un décret est de portée générale. Nous pourrions ajouter, mais j'entends la différence que vous faites entre les départements les plus touchés et les départements qui le seraient moins,

Mme Christine Lavarde. Le Gouvernement a décidé de remettre en place le dispositif de qui avait déjà été utilisé pour faire face aux conséquences de la crise financière de 2008.

mais également le stock de créances déjà constitué. Or, en reprenant la rédaction de l'article 220 en vigueur et en disposant que l'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, vous serez peut-être amenée à restreindre la portée de l'article 2 en excluant

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement vise à élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances consentis aux petites entreprises éligibles au fonds de solidarité. En incitant les créanciers à renoncer aux créances ou loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux petites entreprises de se désendetter et d'aborder la reprise dans de meilleures conditions. Il éviterait par ailleurs à l'État d'absorber le paiement de ces créances ou loyers le fonds de solidarité, ce qui diminuerait de fait le coût pour les finances publiques du soutien aux petites entreprises. En l'état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créances à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu'à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent. Les aides et abandons de créances non motivés par des raisons commerciales ne sont pas déductibles. Quel